Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

La fin du cumul des droits à la formation sur l'ensemble du mandat, le passage d'un calcul des droits en heures à un calcul en euros, la baisse des droits à la formation de 2 000 euros à 700 euros par an, ou encore le maintien de la gestion du système par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en dépit de ses frais de gestion mirobolants faisaient partie des points de tension ayant entraîné la colère de nombreux élus. Fort heureusement, la commission des lois du Sénat a depuis retravaillé en profondeur les ordonnances, trouvant une solution plus équilibrée et respectueuse du droit à la formation des élus. Madame la ministre, vous avez été ouverte aux propositions formulées par le Sénat, et je vous en remercie.

D'autre part, je souhaite attirer votre attention sur la nécessité d'un réel contrôle des agréments et des sous-traitances. Il est bien d'avoir créé une procédure de retrait de l'agrément en cas d'abus et une interdiction des sous-traitances de second rang, mais encore faut-il qu'un réel contrôle du respect des obligations incombant aux organismes soit mis en oeuvre. Car, nous le savons, ce sont majoritairement les abus de certains organismes de formation qui nous ont forcés à réformer le DIFE, ce dont les élus pâtissent aujourd'hui. Madame la ministre, vous engagez-vous à véritablement contrôler les rapports annuels d'activité des organismes de formation ? Enfin, je souhaite souligner un point qui n'a, me semble-t-il, pas été abordé lors des débats de la semaine passée. Oui, le budget du fonds DIFE était déficitaire et nécessitait d'engager des fonds publics, ce qui justifiait un rééquilibrage. Mais il faut relativiser le coût que la formation des élus représente pour l'État. Car des élus bien formés, ce sont des politiques locales vertueuses sur le long terme, ainsi que des investissements bien choisis et utiles. Et ce sont aussi des recours contre des décisions des collectivités, donc des frais judiciaires,

Loin de fragiliser le droit à la formation des élus, la réforme le conforte dans tous ses aspects, qu'il s'agisse des dispositifs de financement, de l'accès à l'offre de formation ou de la qualité des formations délivrées.

de contribuer à la formation des conseillers municipaux selon des modalités très souples, sans pour autant prendre la compétence. Cela répondra notamment au besoin de soutien des petites communes, qui peinent à faire face aux demandes des élus.

la responsabilité qui est la nôtre. Il faut effectivement changer de système pour éviter les dérives de certains organismes de formation indélicats ayant conduit

de le remplacer. Le Territoire de Belfort profite depuis le mois de mars 2017 du nouvel hôpital Nord Franche-Comté. Pour répondre à des critères d'accessibilité et de proximité, le choix a été fait d'implanter le site sur la commune de Trévenans, qui compte 1 300 habitants seulement. Or, comme vous le savez, l'installation d'un site hospitalier de cette importance a des conséquences sur la vie de la commune qui l'accueille. Celle-ci doit en particulier comptabiliser les naissances et les décès et supporter en conséquence les frais de gestion de l'état civil,

Une partie des frais restent cependant supportés uniquement par la commune d'implantation. Très concrètement, qu'est-ce que cela implique pour notre petite commune rurale ? En 2020, le coût de fonctionnement du service de l'état civil était de 190 000 euros, euros, dont 62 % seulement étaient récupérables, car des communes extérieures n'atteignaient pas les seuils légaux de 1 % de naissance ou de décès. Résultat : 72 000 euros sont restés à la charge de la commune de Trévenans.

suivant le même principe que l'aide apportée aux communes réalisant les cartes d'identité ou les passeports. Madame la ministre, quelle solution retenez-vous ou proposez-vous ? La parole est à Mme la ministre.

L'attribution de missions en qualité d'agent de l'État ne s'analyse pas comme un transfert de compétence ; il n'y a donc pas d'accompagnement financier. Juridiquement d'accompagnement financier. Juridiquement parlant, les charges d'état civil supportées par la commune de Trévenans ne peuvent pas être compensées par l'État. Toutefois, afin de répondre aux situations exceptionnelles, la loi a prévu le principe d'une répartition des dépenses d'état civil au profit d'une commune ayant sur son territoire un établissement de santé accueillant un public provenant de l'extérieur. Ce mécanisme se traduit par une contribution financière des communes extérieures, qui repose- vous l'avez souligné -sur la différence entre les naissances comptabilisées au sein de l'établissement et le nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement de santé. Une contribution financière s'applique s'applique à toutes les communes ayant plus de 1 % de naissances ou de décès dans l'établissement. Il revient ensuite aux élus de s'organiser pour se mettre d'accord sur leurs contributions respectives. Ils peuvent aussi créer un service commun (EPCI) et ses communes membres, afin de mutualiser les charges liées aux missions d'état civil. À défaut d'accord, la contribution de chaque commune est fixée par le préfet.

accessible seulement une quinzaine de jours, alors que les dossiers étaient à déposer entre le 4 janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Plus de 14 000 dossiers ont été déposés, principalement pour du matériel d'épandage et de pulvérisation, excluant de nombreux agriculteurs du dispositif.

-et peut-être aussi un manque de sélectivité des matériels éligibles, suscitant frustrations et incompréhensions. Par ailleurs, les prix de vente des matériels auraient augmenté de 4 % à 15 %. Si cette augmentation est avérée, des contrôles ont-ils été opérés par FranceAgriMer ? ? En outre, les chartes départementales de protection des riverains ont été rendues caduques par une récente décision du Conseil constitutionnel. Alors que débutent les périodes de traitement, l'ensemble de la profession a besoin de sécurité juridique, notamment à la veille de l'ouverture des déclarations de demandes d'aides de la politique Force est de constater que le dispositif d'aide à la conversion aux agroéquipements témoigne de l'engagement de l'agriculture dans la transition agroécologique. Monsieur le ministre, envisagez-vous de nouveaux crédits dans le cadre du plan de relance national ? Quelles sont les réponses juridiques envisagées concernant les chartes avec les riverains ?

nous comptons sur vous et sur le Gouvernement pour activer très rapidement tous les leviers d'accompagnement et mettre en place un plan d'aide et de sauvetage

en place non seulement les dispositifs habituels, mais également des dispositifs exceptionnels- le Premier ministre s'y est engagé -face à cet épisode absolument dramatique. Le problème du gel est qu'il est invisible.

jour ... Ma démarche est relayée par les agriculteurs, et un certain nombre de mes collègues ont cosigné une proposition de résolution en ce sens.

Elle doit permettre aux citoyens de connaître les femmes et les hommes passionnés qui nourrissent la population. Il s'agira d'un geste fort, qui sortira le secteur agricole de son sentiment de découragement et marquera la considération que l'ensemble du pays doit apporter à ses paysans.

et une contribution au PIB de 6,7 %. Notre agriculture est bien la meilleure du monde

les acteurs de la filière font face à une distorsion de concurrence avec nos voisins européens, en particulier sur la protection phytosanitaire du riz et sur le désherbage. Bien Bien que les autorités compétentes sur le sujet aient été plusieurs fois alertées, la situation n'a malheureusement guère évolué, laissant les riziculteurs aujourd'hui dans une impasse technique pour désherber correctement leurs rizières. Ces difficultés entraînent une baisse constante des rendements, mais également des surfaces rizicoles, dont l'étendue se situe désormais au-dessous de 15 000 hectares alors que 20 000 hectares étaient cultivés voilà une dizaine d'années. La sole riz 2021 est, à titre d'exemple, estimée à 8 000 hectares. En outre, cette diminution du volume de culture a des conséquences dramatiques sur le paysage et la biodiversité camarguaise. L'important apport en eau douce nécessaire à la riziculture a vocation à irriguer toute la nature environnante. En effet, en présence de la nappe phréatique extrêmement salée de ce territoire, la submersion régulière des parcelles grâce au riz est indispensable pour permettre à la terre de ne pas devenir stérile à cause de trop grandes remontées de sel. Monsieur le ministre, pouvons-nous à cet égard compter sur votre aide pour harmoniser les moyens de production de nos riziculteurs avec nos voisins européens, afin que la riziculture française, indissociable de l'identité de la Camargue, au même titre que l'élevage de taureaux et de chevaux Camargue, puisse envisager l'avenir avec sérénité ? Bravo ! La parole

une évolution du protocole vaccinal aux éleveurs. Pour les broutards, ils disposent d'un délai de soixante jours, contre dix jours jusqu'à présent, entre la date de la dernière injection de vaccin et la date de la vente pour l'exportation. Pour les animaux dont la vente est programmée en avril 2021, il fallait donc avoir réalisé tout le protocole vaccinal au plus tard le 30 janvier 2021, une date évidemment impossible à tenir. Or près de 6 200 broutards devraient être exportés en avril et en mai pour le seul département de la Haute-Vienne. En l'absence d'une telle opération réalisée dans les temps, ces ventes ne pourront donc pas être conclues, et on mesure aisément la perte pour des producteurs déjà en grande difficulté. Il semblerait que la situation n'ait pu être anticipée, et la légitime demande des éleveurs pour l'obtention d'un temps d'adaptation à ce nouveau règlement européen n'a pas été entendue. Monsieur le ministre, quelle mesure de compensation avez-vous donc prévue pour les dédommager ? Cette situation est d'autant plus préjudiciable que la filière bovine limousine fait déjà face à une baisse des cours, en raison de fortes perturbations sur les marchés européens liées au contexte sanitaire. Si les exportations de broutards et de jeunes bovins vers l'Italie restent stables, le prix payé au producteur est en baisse :-3 % sur toute la voie mâle, et un écart d'environ 1 euro au kilogramme entre le prix payé au producteur et l'indicateur interprofessionnel de coûts de production. Cette baisse de prix annule tout le gain de revenu potentiel qu'aurait pu procurer la hausse de 40 centimes du kilogramme obtenue sur la voie femelle, entraînant de fait un

Ce n'est absolument pas le cas. Vous pouvez d'ailleurs interroger les représentants de la filière à cet égard. Le fait est que la France s'est battue au niveau européen pour que cette réglementation n'entre pas en vigueur au 21 avril, mais soit décalée. J'en ai parlé à de nombreuses reprises ; j'ai fait une coalition avec différents États membres

la date du 21 avril de manière sereine, puisqu'il y aura une autre échéance au mois de septembre, avec des protocoles d'accord sur les vaccinations pour les exportations,

d'autant que, depuis 2018, le revenu des éleveurs bovins « viande » a baissé de 30 %. Les ventes de viande bovine, elles, ont progressé en 2020, mais le problème est bien que la loi Égalim n'est pas appliquée et n'a pas produit les effets positifs attendus. Les plans d'aide d'urgence successifs, tels que celui qui a été annoncé début mars, ne suffisent plus à répondre à cette situation. Il faut garantir aux éleveurs un prix qui couvre véritablement leurs coûts de production. La nouvelle PAC ne doit pas sacrifier l'élevage allaitant, sous peine de porter gravement atteinte aux équilibres territoriaux et à notre autonomie alimentaire.

Un profond désaccord entre les parties s'est traduit par des manifestations d'agriculteurs partout en France, ces derniers dénonçant la teneur de ces négociations et demandant une application de la loi Égalim beaucoup plus juste. Le problème est bien là ! Rappelons

Ils ont le sentiment que la grande distribution est peu réceptive aux tarifs proposés par les fournisseurs et que la hausse des coûts de production à l'amont n'est absolument pas prise en compte. D'ailleurs, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ne dit pas autre chose quand il affirme que, dans de très nombreuses filières, les prix payés aux producteurs n'intègrent pas suffisamment les coûts de production. Monsieur le ministre, la crise sanitaire a mis en avant l'importance stratégique de préserver notre souveraineté alimentaire. Cela passe, vous le savez, par une juste rémunération de nos agriculteurs, leur permettant de répondre aux exigences sociétales et environnementales de plus en plus contraignantes.

en nombre. Allez-vous vous saisir du rapport de Serge Papin pour mieux rémunérer les agriculteurs ? Plus globalement, quelles mesures comptez-vous prendre pour que la rémunération des agriculteurs reflète réellement leur travail ?

est envisagée à l'heure actuelle, équivaudrait à près de 180 millions d'euros par an d'aides en moins. C'est colossal et, vous le comprendrez, inacceptable. Nos agriculteurs ont plusieurs ont plusieurs propositions à vous faire sur le plan stratégique national, en cours d'élaboration. Je vous demande, monsieur le ministre, de les écouter. Nous ne devons pas avoir honte de soutenir notre agriculture. monsieur le ministre,

Malgré les très nombreuses interpellations et propositions des syndicats agricoles depuis deux ans, les mesures de biosécurité déployées pour protéger les élevages des maladies ont essentiellement été envisagées pour des élevages intensifs et paraissent largement inadaptées à la réalité des élevages extensifs. C'est encore plus le cas dans les territoires de montagne comme le mien. Depuis le 1 janvier, les éleveurs porcins attendent des dérogations, notamment sur la question des clôtures. Les systèmes de clôture pour les parcs à cochons ne sont pas adaptés et peuvent conduire à l'arrêt de l'élevage porcin extensif, particulièrement en zone boisée ou pentue. (Anses) a enfin été saisie et doit se prononcer sur la possibilité de déployer des clôtures mobiles, beaucoup plus adaptées à l'élevage de plein air. Monsieur le ministre, savez-vous quand l'Anses rendra son rapport ? Cette situation est d'autant plus mal vécue par les fermes de plein air qu'aucune nouvelle réglementation sanitaire ne s'impose aux chasseurs,

S'agissant de la grippe aviaire, à la suite de la pétition de cet hiver, vous avez réuni depuis mars les acteurs pour élaborer un protocole adapté à tous les types d'élevage. Nous attendons de voir le résultat, résultat, mais, enfin, claustrer les volailles pour les protéger de la grippe aviaire dans des bâtiments construits avec les subsides du plan de relance ne me semble pas être une solution pour l'élevage de plein air. Je m'étonne de devoir le préciser. Plus largement, monsieur le ministre, que prévoyez-vous pour protéger et développer l'élevage de plein air

ma question porte sur les conséquences de l'arrêt des exportations de laine française à la suite de la crise sanitaire, ainsi que sur les perspectives de renaissance de la filière de production et de valorisation de la laine sur notre territoire. La France possède un cheptel de près de 5 millions de brebis, qui produisent un peu plus de 6 000 tonnes de laine par an. Depuis des décennies, la filière de production de la laine tricolore a chuté. On élève surtout les ovins pour la viande ou le lait. La vente des tontes suffit à peine à en payer l'acte actuellement. C'est pourtant malheureusement un passage obligatoire pour le confort de l'animal et pour lutter contre la myiase. Notre production de laine s'exporte à hauteur de 80 %, principalement vers l'Asie. Or, depuis la crise de la covid-19, la Chine a coupé court à ses importations et les stocks s'accumulent de manière alarmante dans les hangars de nos éleveurs.

S'ils demeurent en l'état, il faudra trouver une solution pour s'en débarrasser. Sans accompagnement, et en l'absence de règles et de contrôles, les éleveurs seront contraints de faire le travail de destruction eux-mêmes, avec toutes les conséquences économiques et sanitaires

que ce soit de Business France ou des conseillers agricoles. Enfin, au-delà de la filière et de ses débouchés, je crois beaucoup aux initiatives locales, telles que celles que vous avez mentionnées. C'est exactement la même approche que pour la valorisation des circuits courts dans le cadre des projets alimentaires territoriaux. Ces valorisations locales sont, à mes yeux, extrêmement importantes. Vous avez cité plusieurs initiatives, et il faut les soutenir.

Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur trois points. Tout d'abord, il y a la prise en compte de la différence « montagne » dans le futur plan stratégique national. Nous constatons que l'éligibilité des surfaces pastorales sera subordonnée à une méthode de déclaration et de contrôle qui reste en débat. L'actuelle repose sur l'expertise de l'agriculteur, qui applique une classe de prorata aux surfaces qu'il déclare. Cette méthode a fait ses preuves en France, mais elle est aujourd'hui en évolution, et je crois savoir que vous expérimentez à ce jour un dispositif de télédétection en vigueur chez nos voisins espagnols et dénommé le Lidar. Il s'agit d'une technique de mesure à distance capable d'identifier le couvert végétal en place. Certes, ce système paraît simple, mais son utilisation est limitée, car il exclut systématiquement toute surface en pente ou toute ressource fourragère sous couvert arboré. L'Association nationale des élus de la montagne (ANEM), notamment, a manifesté son opposition à cette nouvelle méthode. Comment allez-vous prendre en compte les spécificités géographiques des surfaces agricoles montagnardes ? Ne pensez-vous pas qu'une dérogation soit nécessaire pour les territoires de montagne ? Ensuite, en cette période d'actualité singulière, avec les gels sévères que connaît le territoire national, j'ai pris acte avec beaucoup de satisfaction de la prise en compte rapide des calamités agricoles. Cela étant, je souhaiterais connaître les dispositions que vous envisagez de prendre pour faire face immédiatement aux besoins de trésorerie auxquels seront confrontés les exploitants arboricoles dès le mois d'octobre, après que les premières recettes des saisons précédentes auront été effectivement liquidées. J'aimerais également savoir quelles mesures vous envisagez

Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions. Je vous invite dans mon département, dans la vallée de la Durance et le Buëch, afin que vous puissiez vous rendre compte de la situation, même si je sais que vous en êtes conscient. Nous pourrons à l'occasion aussi parler de pastoralisme.

sur les conséquences importantes, pour le service public d'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Roanne, que risquent d'entraîner les nouvelles réglementations relatives aux conditions de retour au sol des boues d'épuration urbaines. En effet, les 10 000 tonnes produites chaque année par les 35 stations d'épuration de ce territoire font l'objet d'une valorisation agricole dans le cadre de plans d'épandage, pour 50 %, et sous la forme de compost, pour 50 %. Or le projet de décret relatif aux critères de qualité agronomique et d'innocuité selon les conditions d'usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture prévoit l'interdiction, à compter du 1 juillet 2021, de tout épandage de boues urbaines non hygiénisées. Par ailleurs, ce même projet de décret, ainsi que celui qui est relatif au compostage des boues d'épuration et digestats de boues d'épuration avec des structurants vont également imposer de très fortes contraintes sur la fabrication et la distribution des composts. Toutes ces dispositions vont entraîner d'importants surcoûts pour leurs services d'assainissement. Soit ces surcoûts seront répercutés sur les redevances d'assainissement payées par les usagers, soit ils seront amortis par une baisse drastique des programmes d'investissement. Au-delà de cette question financière cruciale, l'agglomération de Roanne et son prestataire de compostage ne pourront pas répondre à ces nouvelles exigences dans les délais prévus, car ils ne possèdent ni les équipements ni les infrastructures nécessaires

En conséquence, madame la secrétaire d'État, je vous demande de bien vouloir prendre en compte toutes les difficultés que posent ces nouvelles réglementations, de les limiter aux exigences strictement nécessaires et de prévoir des délais compatibles

Ces normes trouvent leur fondement dans l'article 86 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui est de fait assez exigeante quant au niveau d'innocuité à atteindre pour permettre le retour au sol de ces boues. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, responsable de l'élaboration des normes de qualité des matières

pour avis au Conseil d'État. Je tiens enfin à vous signaler que des moyens ont été mis en place dans le cadre de France Relance : une enveloppe de 30 millions d'euros d'aide d'urgence vient aider les collectivités à

je souhaiterais vous interpeller sur le financement de l'objectif « zéro artificialisation nette », qui est l'une des grandes thématiques du projet de loi Climat et résilience. L'article 47 de ce projet de loi dispose que le rythme de la consommation foncière doit être divisé par deux d'ici à 2030 ; son article 48 précise que l'action des collectivités doit limiter l'artificialisation des sols. L'objectif est certes louable et les élus sont conscients de la nécessité de réduire le plus possible les consommations foncières et l'artificialisation ; toutefois, ils s'interrogent sur le modèle de financement et les modalités concrètes d'application L'objectif est national, mais ce sont les élus locaux qui vont être à la manoeuvre en matière d'urbanisme ; or les inquiétudes sont nombreuses. Votre projet de loi invite principalement à modifier les documents d'urbanisme- plans locaux cela n'est pas suffisant. Le projet de loi fixe la ligne directrice, mais il ne donne pas aux collectivités les outils et les moyens pour y parvenir. Sur le principe, la majorité des élus est d'accord, mais concrètement, on ne sait pas comment y arriver

Ma question est donc simple : concrètement, quel est le mode d'emploi de l'objectif « zéro artificialisation nette » ? Comment financer cet objectif ? Quels sont les leviers, notamment fiscaux, prévus pour les collectivités ? La parole est à

conformément à la recommandation de la Convention citoyenne pour le climat. Chaque année, entre 20 000 et 30 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers sont artificialisés, avec des conséquences écologiques que personne ne nie, mais aussi des conséquences socioéconomiques, telles que la dévitalisation des petites centralités, l'éloignement de l'emploi et des surcoûts pour la Je partage donc votre analyse : l'un des principaux moteurs de l'artificialisation des sols est bien économique. En effet, il est

Le différentiel de coûts est d'autant plus élevé lorsque les opérations se situent sur des friches et dans des secteurs détendus, qui ne permettent pas de générer des recettes pour équilibrer le bilan économique de l'aménagement.

Aussi, afin d'apporter des réponses en matière de financement du « zéro artificialisation nette », le ministère de la transition écologique envisage trois leviers principaux. Le premier levier est le développement de l'ingénierie foncière et financière des établissements publics fonciers (EPF), qui acquièrent du foncier, le remettent en état et le gardiennent avant rachat à prix coûtant à la collectivité dans le cadre d'une convention. Leur modèle économique repose sur la recette fiscale de la taxe spéciale d'équipement. Cette taxe est votée dans les conseils d'administration des EPF, qui sont toujours présidés

Comme trop souvent, le Gouvernement se borne à fixer de grands principes et des objectifs, sans considérer leurs aspects opérationnels. En fonctionnant ainsi, l'État prend uniquement une position de contrôle ; cette défiance est mal perçue sur le terrain. Je vous invite donc à ne pas vous précipiter et à travailler en concertation avec les collectivités et les élus locaux, afin d'aboutir à un véritable mode d'emploi pour la mise en oeuvre de cet objectif. La parole est à M. Laurent Burgoa,

À l'heure où la conscience écologique s'éveille chaque jour un peu plus, cette situation est de moins en moins compréhensible. Il manque à la gare de Nîmes-Pont-du-Gard une troisième voie propre à assurer des correspondances adaptées aux cadencements des TGV. Pourtant, les moyens financiers sont quasiment réunis pour satisfaire

Ainsi, sollicité par les collectivités partenaires- communauté d'agglomération, département du Gard et région Occitanie -, le préfet de région a saisi SNCF Réseau, il y a plusieurs mois, en vue de la préparation d'un ultime comité de pilotage. Or le représentant de l'État et les collectivités cofinanceuses s'entendent répondre par SNCF Réseau que ses services ne sont toujours pas en mesure de fournir le bilan comptable de l'opération, qui préciserait le montant exact du reliquat, ce qui repousse toute Enfin, si le soutien de la région comme du conseil départemental au principe de l'affectation intégrale de cette somme à la troisième voie a été clairement exprimé, il n'en demeure pas moins que l'immobilisme de SNCF Réseau est préjudiciable au développement touristique et économique de notre territoire. comme vous l'aurez compris, je vous demande de bien vouloir user de toute votre autorité pour que SNCF Réseau rende des comptes, au sens propre comme au sens figuré, dans les plus brefs délais ! Oui, cela s'impose, car il est aberrant de devoir compter sur le bus ou la voiture pour se rendre à cette gare. La parole

Burgoa, vous nous interrogez à propos des dessertes ferroviaires de la gare de Nîmes-Pont-du-Gard. Comme vous le rappelez, les élus nîmois ont exprimé le souhait que soit créée, sur la ligne classique, une troisième voie à quai permettant l'organisation de navettes TER entre la gare nouvelle et la gare centrale de Nîmes. Dans cette optique, ces navettes TER relieraient les deux gares en huit minutes, la troisième voie permettant à la navette de stationner en gare nouvelle dans l'attente du passage des TGV.

opération. À ce stade, le conseil régional d'Occitanie, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, s'est plutôt engagé dans le cadre de la nouvelle convention TER en faveur de l'arrêt systématique de 44 TER en gare nouvelle, plutôt que de la réalisation d'une navette ferroviaire dédiée en dehors du réseau. Ce sujet recevra en

À terme, en desservant dix gares entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes, cette ligne traversera un bassin de vie de 700 000 habitants et de 300 000 emplois. Devant ces chiffres, vous imaginez aisément l'attente légitime que cette réouverture suscite au sein de la population. Porté et financé par la région Occitanie, ce projet devait initialement aboutir à une mise en service en décembre 2021. Cela avait été acté lors des différents échanges entre la région et SNCF Réseau.

tout un arsenal de procédures, ce qui ne permettrait pas d'envisager une réouverture de la ligne aux passagers avant 2023. Ces procédures complémentaires sont pertinentes et logiquement prévues dans le cadre d'une ouverture de ligne. Pour autant, au moment où je parle, la ligne de la rive droite du Rhône voit déjà circuler quotidiennement des trains de fret et même occasionnellement des TGV, qui l'utilisent comme itinéraire de substitution.

à l'heure où la transition énergétique est à la fois un impératif et une urgence, pouvons-nous nous permettre de retarder un tel projet ? Aussi, compte tenu de ces éléments, le Gouvernement compte-t-il intervenir afin de lever les obstacles qui s'opposent encore à une réouverture rapide de la ligne de la rive droite du Rhône aux passagers ? La parole

Cependant, des TER circulent sur la section Avignon-Nîmes, sans arrêts intermédiaires ; la voie sert également d'itinéraire de détournement pour la ligne de la rive gauche. Elle reste parcourue par environ vingt trains de fret par jour et fait partie d'un corridor européen. La région Occitanie porte un projet de reprise des TER entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit ; on desservirait ainsi dix gares, dont huit doivent être remises en exploitation, pour huit allers-retours quotidiens. La mise en service complète de cette pour le service annuel 2026, mais la région a souhaité prévoir une première phase dès la fin de l'année 2021. Cette échéance avancée est néanmoins apparue difficile à tenir, compte tenu d'un certain nombre de règles de sécurité ferroviaire dont personne ne souhaite, à l'évidence, s'affranchir trop rapidement ; il convient de les respecter dès qu'il qu'il y a renouvellement ou réaménagement d'une ligne. La sécurité des passages à niveau fait notamment l'objet d'une forte attention. L'ampleur du projet et le nombre de passages à niveau ont conduit l'Établissement public de sécurité ferroviaire à demander en décembre 2020, comme vous l'avez rappelé, la production d'un certain nombre d'études nécessaires pour délivrer les autorisations réglementaires.

différente de la manière dont vous envisagez la mise en oeuvre concrète de la séquence dite « ERC »- éviter, réduire, compenser -, qui est au coeur du processus d'évaluation environnementale de tout projet, depuis sa conception et pendant toute sa durée de vie. de vie. Les mesures compensatoires ne sont actuellement pas garanties, alors qu'elles font l'objet d'une obligation de résultat dont les maîtres d'ouvrage sont débiteurs. Pour toutes ces raisons, je regrette les atermoiements récurrents autour de ce dossier que nous portons auprès du Gouvernement depuis 2018. À ce titre, je réitère ma volonté d'être reçu, ainsi que mes collègues parlementaires cosignataires de ce courrier, par M. Djebbari ou ses services. Des solutions existent, notamment en matière de protection phonique. Nous nous devons de les faire émerger le plus rapidement possible pour l'ensemble des riverains de ces lignes, qui sont quotidiennement confrontés à des nuisances sonores. La parole

Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. Ensuite, nous travaillons sur les normes et la qualification du bruit. Quand ces nuisances sont avérées, en dépit du respect global de la réglementation, elles seraient liées non pas à un niveau de bruit régulier, mais à des pics de bruit élevé lors du passage des trains. Sur ce deuxième point, les travaux se poursuivent, en lien notamment avec l'arrêté du 8 novembre 1999

être menées et un consensus final doit être recherché. Ces travaux permettront d'enrichir les connaissances et d'améliorer les pratiques en matière d'évitement, de réduction et de compensation des impacts, la fameuse séquence ERC

l'Association des familles victimes du saturnisme nous a alertés sur le risque d'intoxication par le plomb des enfants vivant dans des logements anciens et dégradés. Les lacunes de la réglementation actuelle relative au constat ne s'applique qu'aux logements construits avant 1949 ; or les peintures au plomb ont été commercialisées jusqu'en 1993. Une étude menée entre 2008 et 2014 a mis en évidence la présence de plomb dans la moitié des logements construits avant 1949 22 % des logements construits entre 1949 et 1974. Aussi, le CREP devrait être étendu au moins aux logements construits jusqu'en 1974. Par ailleurs, l'intoxication au plomb par l'eau du robinet

dans certains sols autrefois affectés à l'épandage d'eaux polluées, mais aujourd'hui potentiellement cultivés, ou affectés à des aires de jeux. Enfin, les crèches et les écoles ne sont pas soumises à l'obligation de délivrance d'un CREP, étant donné que ce dernier ne concerne que les bâtiments destinés à un usage d'habitation. Aussi, nous devons devons veiller à étendre le dispositif de prévention. Le saturnisme est une maladie qui touche surtout les enfants des quartiers défavorisés et ceux qui vivent dans des logements en mauvais état. Il comporte des risques graves pour les jeunes enfants et peut causer une atteinte irréversible des facultés cognitives. Les cas de saturnisme sont encore trop nombreux en France et les dépistages restent insuffisants. Madame la secrétaire d'État, au regard de ces différents éléments, une mise à jour de la réglementation relative à la prévention du risque d'intoxication au plomb semble nécessaire. Quelle suite entendez-vous donner à cette demande ? La parole est à Mme la secrétaire

prennent particulièrement en compte les risques liés à la fréquentation par un enfant d'un logement ou d'un bâtiment- notamment une crèche ou une école -construit avant 1975, et non avant 1949, et dont les peintures seraient écaillées. Cela concerne également les logements qui comportent des canalisations en plomb. S'agissant de la réglementation actuelle concernant les constats de risque d'exposition au plomb, l'arrêté du 19 août 2011 s'inscrit dans une logique de prévention primaire du risque saturnin : il s'agit bien d'identifier les logements à risque pour pour que la réalisation de travaux supprime toute accessibilité du plomb. Cette obligation concerne les logements construits avant 1949, année de l'interdiction des peintures contenant de la céruse à très forte concentration en plomb. Les Les bâtiments non destinés à un usage d'habitation, tels que les crèches ou les écoles, ne sont pas soumis à cette obligation. Pour ce qui concerne ces établissements, l'instruction du 21 septembre 2016 contient une incitation à la réalisation de de CREP pour la recherche de sources d'intoxications dans le cadre des enquêtes environnementales autour de cas de saturnisme infantile. Par ailleurs, le risque saturnin est pris en compte dans les polices administratives spéciales de lutte contre l'habitat indigne. Ce dispositif est détaillé dans l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations. Au regard des mesures de santé publique mises en oeuvre et de tous ces éléments, nous prenons bien évidemment en considération vos propositions visant à faire évoluer cette réglementation. Elles seront étudiées en lien avec le ministère chargé du logement.

Bien plus prévisible et antérieure à la covid-19, elle met en tension les services de soin du territoire sarthois. En effet, la désertification médicale dans nos territoires tend à exacerber l'explosion des maladies professionnelles et générales dans les classes populaires. Ces inégalités sociales et de santé sont directement liées à la désertification rurale, entraînant de fait une exposition plus sévère au virus des populations les plus fragiles. En 2019, un homme de milieu rural vit en moyenne 2,2 années de moins qu'un hyperurbain. L'écart est de 6 ans entre un ouvrier et un cadre. C'est pourquoi la revitalisation de services publics hospitaliers performants dans nos territoires est un enjeu tant de santé publique que de justice sociale. À ce titre, j'attire votre attention sur le centre hospitalier de Montval-sur-Loir, dans la Sarthe. Ce centre hospitalier compte parmi les sept établissements hospitaliers du département sarthois, lequel est déjà durement touché par la pénurie de personnel médical et paramédical depuis des années. années. Ainsi, en 2015, un arrêté ministériel a classé comme « isolé » ce service des urgences. Depuis la mi-2019, le service des urgences a connu des fermetures temporaires régulières, faute de personnel. La situation du service des urgences a inévitablement des conséquences sur le service d'hospitalisation complète de médecine, car la quasi-totalité des séjours de médecine se fait par les urgences. Alors que les pathologies psychiques explosent en ces temps de confinement, cet hôpital accueille un centre médico-psychologique ainsi que les consultations de pédopsychiatrie. L'hôpital se situe dans un département où la démographie médicale constitue un enjeu majeur. Plus de 40 000 Sarthois sont sans médecin traitant et l'érosion du nombre de praticiens devrait encore s'accentuer dans les prochaines années. Madame la ministre, je tiens à porter à votre attention le fait que cet établissement périclitera tant que les autorités publiques de santé ne mettront pas d'importants moyens pour en assurer la pérennité. La crise sanitaire que notre pays traverse nous rappelle l'impérieux besoin d'investissements matériaux et humains dont l'hôpital public a tant besoin. Ce qui n'était pas envisageable avant la covid-19 devient impératif aujourd'hui.

Ce service d'urgence accueille un peu plus de 8 000 patients à l'année et connaît depuis plusieurs mois, comme vous le soulignez, de très fortes tensions de professionnels de santé, notamment de médecins urgentistes. Les départs de médecins de ce service et les difficultés récurrentes de recrutement expliquent les fermetures temporaires mais régulières du service des urgences et le tableau de gardes incomplet par moment.

(GHT). Est également mené avec l'université d'Angers un travail visant à orienter des médecins juniors vers le service d'urgence du Mans pour soutenir Montval-sur-Loir. La recherche de médecins est très active, y compris au sein des établissements publics du département et de la région. Par ailleurs, cet établissement bénéficiera, en 2021, du label « hôpital de proximité », donc d'un soutien et d'un accompagnement financier constants l'ARS Pays de la Loire. Près de 350 000 euros ont été accordés pour rénover le plateau des consultations et acquérir un échographe. L'ARS accompagnera aussi, en investissement d'amorce, la rénovation du service de soins de suite et de réadaptation, à hauteur de 350 000 euros supplémentaires pour améliorer la qualité et l'attractivité professionnelle territoriale. Monsieur le sénateur, le 25 février dernier, avec le soutien du ministère, le directeur de l'ARS et la présidente du conseil régional se sont rendus sur site pour réaffirmer l'importance de cet établissement de proximité que nous suivons avec grande attention.

C'est l'expression de la solidarité nationale, que je partage avec vous. À cette fin, la caisse nationale d'assurance maladie doit évidemment mobiliser tous les moyens disponibles pour être en phase avec les besoins de l'ensemble de ses publics et s'adapter. À cet égard, l'accueil physique demeure un canal de contact privilégié, notamment pour les assurés en situation de précarité financière. C'est pourquoi l'assurance maladie déploie, dans le département de la Seine-Saint-Denis, un réseau particulièrement dense de quatorze agences. Elle procède à des recrutements supplémentaires d'une trentaine d'agents pour assurer l'accueil des usagers et fait évoluer son tissu d'accueil pour l'adapter. Néanmoins, certains sites anciens, devenus inadaptés aux besoins, sont relocalisés dans des surfaces plus grandes et plus accessibles au regard de l'offre de transports. À titre d'exemple, la CPAM a annoncé l'ouverture prochaine de nouvelles agences à Aubervilliers et Clichy-Sous-Bois, tout en capitalisant sur le déploiement du réseau France Services pour assurer un service supplémentaire de proximité pour les usagers d'autres communes. Pour s'assurer que la reconfiguration des sites d'accueil sur le département s'effectue sans rupture de l'accueil des usagers, le processus a fait et continuera de faire l'objet de concertations avec les collectivités concernées.

d'accueil physique, d'orientation des assurés et, plus généralement, d'accès aux droits et de l'« aller vers ». Ce sont autant de défis que nous devons relever ensemble en nous appuyant sur le partenariat local. Le Gouvernement sera évidemment vigilant pour que la continuité territoriale soit assurée et l'accessibilité garantie dans cette restructuration. Je vous remercie de m'avoir posé cette question qui me permet de le rappeler.

ministre des solidarités et de la santé. Madame la ministre, le 31 mars dernier, le Président de la République a annoncé la création de nouveaux lits de réanimation, afin de mieux faire face à la pandémie de covid-19. Permettez-moi donc d'évoquer le cas de l'hôpital de Beaumont-sur-Oise. En effet, dans le cadre d'un schéma régional de restructuration de l'offre de soins piloté par l'ARS d'Île-de-France, cet établissement a vu, au 1 septembre 2019, le démantèlement de tout ou partie des services de néonatalogie, de réanimation, de chirurgie conventionnelle et de pédiatrie. Cela représente plus de 200 lits et 200 postes de travail, dont 8 lits de réanimation et 4 lits de soins continus. Inutile de dire que ces lits se seraient avérés plus que précieux au coeur de la crise sanitaire dramatique que notre pays traverse. Inutile de dire aussi qu'ils auraient pu éviter des opérations fatigantes et coûteuses de transferts de malades. Inutile de dire, enfin, que la densité du maillage médical est l'une des clés indispensables indispensables à une prise en charge optimale de la santé d'une population. Le triste feuilleton sans fin du covid-19 l'a démontré, s'il en était besoin. Heureusement, une erreur peut toujours être corrigée. Ainsi, la réimplantation d'un service de réanimation à Beaumont-sur-Oise est à la fois possible, souhaitable et souhaitée. Ce réaménagement ne pose, par ailleurs, aucun problème technique, le plateau ainsi que le réseau de fluides étant toujours présents. Le périmètre couvert par cet établissement représentant plus de 180 000 habitants du nord du Val-d'Oise et du sud de l'Oise, il s'agit là d'un enjeu de santé majeur. Aussi, j'espère très sincèrement que la situation du centre hospitalier de Beaumont sera réexaminée avec pragmatisme, objectivité et avec pour seule priorité la protection médicale de la population. De très nombreux élus- je pense notamment à ceux de Méru et Chambly -et habitants de ce territoire, n'ayant pas compris et refusant cette décision unilatérale de l'ARS Île-de-France, sont toujours mobilisés et en attente de ce « réarmement médical ». Madame la ministre, personne ne comprendrait, après les annonces du Président Macron, et alors qu'une solution rapidement opérationnelle s'offre aux pouvoirs publics, que les lits de réanimation de Beaumont-sur-Oise ne soient pas rouverts.

où le système hospitalier est soumis à une pression extrêmement forte. C'est un enjeu de court terme, auquel nous répondons, comme de long terme, pour lequel nous développons des solutions historiques, au moyen du plan d'investissement prévu

ont montré leur formidable capacité à s'adapter très rapidement, avec l'appui des agences régionales de santé, pour faire face à l'épidémie et accueillir en réanimation tous les patients qui devaient l'être. En Île-de-France, se déploient

S'agissant du centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise, il a été décidé, en 2019, de rassembler sur le site de Pontoise les 18 lits de réanimation du centre hospitalier de Pontoise et les 8 lits du centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise, soit 26 au total. Ce regroupement a permis de mieux utiliser les capacités de réanimation de cette partie du Val-d'Oise. Aujourd'hui, le centre hospitalier a déjà ouvert 4 lits de réanimation supplémentaires et soigne donc 30 patients covid en réanimation. l'établissement peut aller encore au-delà si nécessaire. Les soins de réanimation restent des soins très lourds pour des cas graves de covid, dont malheureusement certaines personnes ne réchappent pas. Tout doit être fait pour enrayer la propagation du virus et prévenir les cas de forme grave. Dans le même temps, nous faisons tout pour que l'ensemble de ceux dont l'état de santé le nécessite bénéficient des soins de réanimation dans les conditions de prise en charge habituelles. L'ARS et sa délégation départementale évaluent toutes les options disponibles, en connaissance du territoire, pour capitaliser sur les choix de réorganisation de 2019 avec

La parole est à Mme Sonia de La Provôté, en remplacement de Mme Catherine Morin-Desailly, auteure de la question n°

Cette dynamique positive permet aux jeunes de développer des compétences et une expertise fortement valorisées sur le marché de l'emploi. Depuis les annonces gouvernementales de l'été 2020 sur le soutien à l'apprentissage- pour rappel, une aide au recrutement en faveur des entreprises est de 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans, et de 8 000 euros pour un apprenti majeur -certains centres de formation d'apprentis (CFA) sont saturés, comme dans le Calvados ou en Seine-Maritime. Le plan de relance gouvernemental, bien qu'il ait eu un effet attractif positif, a créé un engorgement des CFA. En outre, le rallongement de trois à six mois du délai pour trouver un contrat d'apprentissage, qui permet aux jeunes de rester plus longtemps en CFA, a eu pour conséquence que les formateurs ne trouvent plus de place pour leurs apprentis.

la volonté du Gouvernement de poursuivre son engagement très fort en faveur de notre jeunesse, de la formation et de l'apprentissage, au travers de l'ensemble des outils que je viens de décrire. La parole est à Mme Sonia de La Provôté, pour la réplique.

a autant d'importance que d'autres voies, telles que la filière générale, dans la formation de la jeunesse de notre pays. La période que nous traversons a montré, s'il en était besoin, à quel point les métiers issus de l'apprentissage sont essentiels pour faire fonctionner notre société.

Ils sont 20 000 à se rendre quotidiennement en Allemagne. La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe ont décidé de réformer le versement des allocations chômage, estimant qu'il revenait non plus au pays de résidence de verser les indemnités, mais au pays employeur. La part des indemnités de chômage totales versées par la France à ses travailleurs frontaliers n'est que de 600 millions d'euros annuels, alors que les salaires rapportent plus de 7 milliards d'euros- c'est tout à fait marginal. Un bras de fer est donc engagé parallèlement à la pandémie de covid-19, à la suite de la mise en place du chômage partiel par les gouvernements allemand et français. Les syndicats des travailleurs frontaliers estiment que la réforme va créer des inégalités

La Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt du 12 juillet 2001, avait clairement précisé, sans rien remettre en cause, que, « lorsque les garanties du pays de résidence sont supérieures aux garanties du pays d'emploi, le pays de résidence doit prendre en charge le complément

au coeur de votre question, est aujourd'hui compétent pour le financement des allocations chômage des travailleurs frontaliers. Cette règle de compétence est à l'origine d'un important déséquilibre financier entre les États membres de l'Union européenne. Le nouveau système proposé par la Commission européenne respecte le principe général selon lequel les travailleurs sont affiliés au régime d'assurance chômage de l'État membre dans lequel ils exercent une activité professionnelle. Ainsi, aux termes du projet de révision de la Commission, qui n'a pas encore abouti, l'État d'activité serait désormais compétent pour prendre en charge les prestations chômage d'un demandeur d'emploi frontalier, au-delà d'une certaine durée d'activité. Cette mesure permettrait une répartition plus équitable de la charge financière entre les États membres. J'entends bien les inquiétudes dont vous avez fait part, notamment celles des travailleurs frontaliers s'agissant des déplacements et des communications qu'imposerait un tel projet.

des conditions de suivi de ces publics. La France est en faveur d'une réforme conciliant la recherche de l'équité financière et des mesures d'accompagnement favorables pour les travailleurs frontaliers. Vous aurez certainement noté que la proposition de la Commission frontaliers la possibilité de s'inscrire en supplément auprès des services de l'État de résidence, ou d'exporter leurs prestations chômage vers leur pays de résidence. Enfin, nous sommes très attentifs à la question de la double charge fiscale, que vous avez évoquée et qui pèse sur les travailleurs transfrontaliers en raison du mode de calcul de l'indemnité de chômage partiel allemand. À ce sujet, nous sommes engagés dans des discussions avec les autorités allemandes. Je ne peux aujourd'hui vous en donner le résultat, mais soyez assurée, madame la sénatrice, que, lorsque nous serons arrivés au terme de ces échanges, nous en communiquerons le contenu. La parole est à Mme Christine Herzog, pour

percevoir un salaire, sauf- et tel est l'objet de ma question -si persistent les dysfonctionnements récurrents de Pajemploi, plateforme visant à simplifier les formalités administratives pour les parents employeurs qui confient la garde de leurs enfants à une assistante maternelle agréée. Dans la réalité, il est plus question de complications, tant pour l'employeur que pour le salarié. Ainsi les assistantes maternelles dénoncent-elles de nombreuses anomalies techniques et administratives, des piratages du site en ligne, des retards de paiement de salaire ou du versement du complément de libre choix du mode de garde par l'employeur. Il arrive également que des bulletins de salaire soient intervertis entre des salariés de toute la France, la divulgation de données personnelles sur le site Pajemploi. Du côté des employeurs, des décalages entre les perceptions d'aides et les prélèvements de charges entraînent des conséquences graves pour les finances de nombreux ménages. Ces situations inacceptables le sont d'autant plus qu'elles ne sont pas récentes. Les nombreuses questions posées à ce sujet par mes collègues sénateurs et députés, depuis plus d'un an, auraient dû vous interpeller.

d'un enfant. Les anomalies que vous évoquez résultent de la mise en oeuvre, depuis juin 2019, d'une réforme du versement du complément de libre choix du mode de garde, ayant accéléré le circuit de versement des allocations Pajemploi pour 850 000 familles.

très concrètes à même de vous rassurer. Comme vous pouvez le constater, même si nous déplorons ces dysfonctionnements et que nous avons agi avec les administrations concernées pour les résoudre, la plupart d'entre eux découlent en fait d'un processus continu de modernisation d'un dispositif au service des parents, qui,

maître de conférences en mathématiques à l'université Claude-Bernard, située sur le campus de Villeurbanne. Depuis très exactement deux ans, ce professeur reste bloqué en Turquie, son pays natal, où il est parti en vacances au printemps 2019. Disposant d'un titre de séjour en France, Tuna Altinel oeuvre, depuis son arrivée dans notre pays en 1996, à d'importants travaux internationaux en algèbre et au développement de la coopération scientifique entre la France et la Turquie. Il est particulièrement investi dans le réseau Universitaires pour la Paix, collectif qui promeut une résolution pacifique du conflit entre l'État turc et les Kurdes.

Pour autant, les autorités administratives du pays ont obstinément refusé de lui rendre son passeport. J'utilise le passé, car, depuis dix jours, une nouvelle étape vient d'être franchie. Le 2 avril dernier, en effet, Tuna Altinel a été informé d'une décision du tribunal administratif en sa faveur. Une décision pourtant prise dès le 25 janvier dernier ! Aussi, vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d'État, il est difficile de se réjouir et de considérer que

poursuites judiciaires en Turquie. La France continue d'appeler la Turquie à respecter ses engagements internationaux en faveur des libertés fondamentales et du droit de chacun à la libre expression. Elle le

Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers. Le 10 novembre dernier, le Gouvernement a publié un décret aux termes duquel tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France [ ...] doit être légalisé », à moins qu'un engagement international n'en dispose autrement. Il peut s'agir d'une convention bilatérale ou de la convention dite apostille en langage diplomatique. Je me réjouis de la réaffirmation, en droit positif, du principe de légalisation ainsi que de la volonté du Gouvernement de pallier les risques d'insécurité juridique résultant de l'abrogation par mégarde de l'ordonnance royale du mois Cependant, je constate avec inquiétude que la légalisation par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l'État ayant émis les actes publics ne peut désormais être effectuée qu'à titre exceptionnel. L'obligation de s'adresser à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français en résidence dans l'État ayant émis les actes publics risque, selon moi, de complexifier les démarches des ressortissants étrangers établis établis en France. Je crains également que cette obligation n'alourdisse la charge de travail des postes diplomatiques et consulaires français situés dans les pays avec lesquels la France n'est pas liée par un instrument international prévoyant une dispense de légalisation. Il est par ailleurs à craindre que certains États n'appliquent pas le principe de réciprocité. Au regard de ces craintes, monsieur le secrétaire d'État, je souhaite connaître les raisons ayant conduit le Gouvernement à restreindre la possibilité d'effectuer les démarches de légalisation auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire en résidence en France. La parole est

En outre, les règlements européens suppriment toutes les formalités d'authentification des actes publics entre États membres. Quand la légalisation l'acte public étranger est d'abord légalisé par l'autorité compétente de l'État émetteur, dont la signature et la qualité sont ensuite certifiées par l'autorité française. Ce sont en effet les autorités présentes dans le pays où l'acte a été établi qui sont les plus à même de pouvoir attester son authenticité. La légalisation par des consulats étrangers en résidence en France ne serait pas plus rapide : ils ne peuvent détenir tous les spécimens de signature de leurs propres autorités et doivent donc interroger les autorités locales à chaque demande de légalisation, ce qui est source de lenteur. Sur les risques de rétorsion, je comprendrais vos craintes si la pratique de la surlégalisation était isolée et nouvelle, mais ce n'est pas le cas.

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez beaucoup de mérite à répondre au nom du Gouvernement à tant de questions qui ne sont pas toujours proches ni du tourisme, ni des Français de l'étranger, ni de la francophonie. Il faut vous en remercier. Ma question a

entre la nécessaire protection du secret de la défense nationale et l'indispensable devoir de transparence en matière historique.

une opération formelle de déclassification avant toute communication. Cette position n'est pas nouvelle. Elle n'a pas varié. L'instruction n° 1300 du 13 novembre 2020 ne fait que l'expliciter. Je comprends le souci que la déclassification préalable n'entraîne n'entraîne pas de délais importants ou de retards significatifs. C'est pourquoi il a été décidé de permettre aux services d'archives, partout où c'est possible, de procéder à la déclassification des documents couverts par le secret de la défense nationale selon le procédé dit de démarquage au carton jusqu'au dossier de l'année 1970 incluse. La mise en oeuvre de cette décision doit conduire à écourter sensiblement les délais d'attente liés à

Monsieur le secrétaire d'État, toute disposition pratique permettant d'accélérer l'accès aux archives historiques est évidemment la bienvenue.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale, ou Dasen, peut ainsi autoriser des dérogations permettant de répartir les enseignements sur huit demi-journées par semaine, alors que, réglementairement, la semaine scolaire comporte vingt heures d'enseignement réparties sur neuf demi-journées. Cependant, selon l'article D. 521-12 du code de l'éducation, ces dérogations ne peuvent pas porter sur une durée supérieure à trois À l'issue de cette période, elles peuvent être renouvelées après un nouvel examen en respectant la même procédure, quand bien même la décision a été prise à la suite d'une consultation des parents. Au cours des dernières années, plusieurs réformes des rythmes scolaires ont touché les collectivités locales. Les équilibres locaux, comprenant parents et enfants, ont besoin de stabilité. De plus, la crise sanitaire complique la réunion des parties prenantes. Madame la secrétaire d'État, dans la mesure où cette dérogation a été prise à la suite d'une consultation des parents, enseignants et élus, seriez-vous favorable à ce qu'elle perdure sans limitation de temps ? Le maire déclencherait de nouveau une consultation si seulement l'une des parties prenantes la réclamait à la suite des trois ans. La parole

que l'étape que nous avons franchie en 2017, conformément aux engagements du Président de la République, a permis de donner davantage de souplesse aux acteurs locaux dans la définition de l'organisation du temps scolaire, afin que

près de 90 % des écoles ont une organisation dérogatoire sur quatre jours, ce qui correspond à environ 85 % des élèves. Conformément à la réglementation en vigueur en matière d'organisation du temps scolaire,

Qu'il s'agisse du cadre général ou du cadre dérogatoire, la décision d'organisation de la semaine scolaire ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. À l'issue de cette période, elle doit de nouveau être arrêtée après un nouvel examen en respectant la même procédure. même procédure. À titre exceptionnel, et parce que la crise sanitaire liée à la covid-19 a rendu plus difficile la réunion des différents acteurs, nous avons permis, par un décret du 25 mai 2020, la prolongation d'un an des autorisations de dérogation

dans la définition des rythmes scolaires, en particulier dans le cadre des OTS dérogatoires. Pour les acteurs locaux, ces concertations constituent une opportunité de réévaluer périodiquement les décisions

Ces troubles envahissants toucheraient plus de 1 % de la population, soit près de 700 000 personnes en France. Les victimes de l'autisme, ce ne sont pas seulement les enfants qui en souffrent, c'est aussi tout leur entourage leur entourage ! Je me suis fortement impliquée à Marseille et au Parlement dans la construction de structures capables d'accompagner l'ensemble des familles. C'est à ce titre qu'est né le projet de l'école Esperanza. Ce projet ne date pas d'hier et me tient particulièrement à coeur, tout comme la construction d'une structure spécialisée pour autistes à l'école Lacordaire, toujours à Marseille, avec la méthode ABA-

c'est le parcours du combattant pour les parents qui se retrouvent souvent dans l'obligation d'arrêter leur travail pour se consacrer avec énergie et amour à leur enfant. Des dispositifs comme Esperanza, médico-éducatif (IME) et l'école inclusive, sont pourtant performants et appréciés des enfants comme des parents. Madame la secrétaire d'État, interpellée par mon collègue député Julien Ravier, vous avez répondu qu'il n'était pas question de fermer les établissements de ce type. Aussi, pouvez-vous nous garantir qu'aucune classe ne fermera ? Dans le cas contraire, quelles sont vos motivations pour désespérer et faire ainsi souffrir les familles et le personnel ?

tous les enfants à 3 ans, y compris ceux qui présentent des troubles plus sévères. La création de 180 UEMA supplémentaires et de 45 unités d'enseignement en élémentaire autisme (UEEA) est ainsi prévue à l'horizon de 2022.

en faveur des élèves porteurs d'un handicap, notamment en faveur de la prise en charge des troubles autistiques. Ainsi, dans le premier degré, 6 nouvelles 6 nouvelles ULIS seront créées, dont 3 spécialisées dans la prise en charge des troubles du spectre autistique (TSA), deux d'entre elles étant situées à Marseille. Le même effort sera réalisé pour les collèges, avec la création de 6 ULIS, dont une ULIS autisme. Enfin, la rentrée 2021 verra dans ce département la création d'une UEMA. Vous le voyez, madame la sénatrice, la rentrée 2021 dans le département des Bouches-du-Rhône, au-delà de la conservation des moyens dévolus à l'école Esperanza, verra une mobilisation significative de moyens supplémentaires en faveur des élèves porteurs d'un handicap. La parole

Agir pour les personnes autistes, c'est conduire un combat pour une vie plus juste, c'est un combat républicain. » Aujourd'hui, votre réponse ne me rassure pas : je veux vraiment savoir si ces quatre classes seront fermées ou non. Vous m'avez garanti les moyens, mais vous ne m'avez pas garanti le maintien de ces classes. J'entends votre plan, mais je sais que les moyens

à nos élèves des soins suffisants et satisfaisants. Pourtant, nous savons qu'un repérage précoce des éventuels troubles de santé est essentiel pour la réussite du parcours scolaire des jeunes enfants. La loi pour une école de la confiance a d'ailleurs prévu, dès la rentrée scolaire 2020, un parcours de santé pour tous les enfants de leur naissance à 6 ans. de leur naissance à 6 ans. Sur le terrain, avec la baisse continue des effectifs de médecins et d'infirmiers, ces objectifs ne sont pas atteints. Selon le Syndicat national des médecins scolaires et universitaires, un médecin scolaire s'occupe en moyenne

La situation est plus grave dans certains départements. Ainsi, dans la Nièvre, département que je représente, sur sept postes de médecins seulement deux sont pourvus. Il manque donc cinq médecins, notamment le médecin conseiller technique auprès de la directrice académique des services de l'éducation nationale. Ce manque a des conséquences lourdes non seulement sur la santé des agents, confrontés à des tâches qu'ils n'assument qu'au prix d'un travail au-delà de leurs capacités, mais surtout sur le suivi médical des élèves. Actuellement, seuls 17 % des enfants de 3 à 4 ans bénéficient d'un examen pour dépister d'éventuels troubles de la vision, de l'audition ou des apprentissages. Les médecins de ville, qui sont déjà en sous-effectifs et surchargés dans bien des territoires, se retrouvent malgré eux à devoir pallier ce manque. Plus largement, l'absence d'une médecine scolaire compromet le nécessaire travail de prévention sur la drogue, les maladies sexuellement transmissibles, la contraception, la nutrition ou encore le harcèlement. En effet, le médecin scolaire est souvent avec l'infirmière le seul

la secrétaire d'État, pourriez-vous me fournir un état des lieux chiffré de la médecine scolaire, à l'échelle nationale et départementale, m'indiquer les mesures envisagées pour doter l'éducation nationale des capacités et des personnels en nombre suffisant ainsi que les délais de mise en place de ces mesures ?

tout d'abord la création de la formation spécialisée transversale de médecine scolaire. Cette surspécialité médicale pour les pédiatres, les généralistes et les médecins de santé publique donne aux étudiants une meilleure connaissance de la profession de médecin scolaire et devrait à terme favoriser le recrutement. Dans la même perspective, des stages de formation de six mois à destination des internes leur sont proposés. Des efforts ont également été réalisés pour doter les médecins scolaires d'outils professionnels numériques plus performants : le déploiement depuis deux ans de l'application professionnelle Esculape, le dossier médical numérique de l'élève, illustre les évolutions des pratiques professionnelles.

Pour mémoire, et parce que c'est toujours un plaisir pour moi de faire référence à son action, mon prédécesseur Michel Raison a déjà sollicité l'analyse du ministère de l'éducation nationale sur ont alors répondu qu'il était prématuré, après une seule année de fonctionnement, de tirer les enseignements de l'expérimentation menée à Jussey. Cette réponse pleine de sagesse était toutefois emplie d'un optimisme communicatif. Elle reconnaissait en effet explicitement l'intérêt du dispositif pour les élèves en milieu rural et l'optimisation de leurs chances de réussite dans ce cadre singulier. Elle soulignait également les efforts déployés par le corps enseignant pour améliorer la continuité des parcours des élèves et des apprentissages. Fort de ces signes positifs, et alors que ce type d'établissement répond à un besoin clairement identifié par certaines collectivités, ma question est somme toute prévisible et logique : quand et comment prévoyez-vous de consacrer les écoles dites du socle ? La

L'organisation pédagogique choisie, qui vise à réunir sur un même site, dans un pôle scolaire unique, des élèves de la petite section de maternelle à la classe de est soutenue par les autorités du département et suivie par les services départementaux de l'éducation nationale. Une attention est portée sur les effets de cette organisation sur la réussite et le parcours scolaires des élèves. Le rapprochement effectif de l'école de la commune de Jussey et du collège au sein d'une même structure bâtimentaire est en cours, et l'ouverture est bien prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2021. Plusieurs temps d'échanges entre les collectivités territoriales compétentes pour chaque niveau scolaire et les équipes pédagogiques concernées ont permis d'aboutir à une réflexion partagée sur les conditions d'accueil à réunir et les choix à effectuer, notamment en matière architecturale, afin d'améliorer la qualité de vie et les conditions d'apprentissage des élèves. Comme vous le savez, la crise sanitaire de la covid-19 et le respect du protocole sanitaire ont eu pour conséquence la suspension de certaines modalités d'organisation et l'impossibilité d'objectiver les effets du projet sur la scolarité des élèves en 2019-2020

des acquis diminue, tant en français qu'en mathématiques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. De plus, on note que la prise en charge de la difficulté scolaire tout au long du parcours des élèves est bien installée dans l'établissement et qu'une amélioration des résultats au diplôme national du brevet (DNB) est perceptible depuis trois ans. outre, les élèves semblent mieux comprendre et vivre les transitions inhérentes au parcours scolaire. Enfin, la création par voie réglementaire ou législative d'établissements publics locaux des savoirs fondamentaux,

les résultats au bout de trois années d'expérimentation, même un peu contrariées du fait de la situation sanitaire, sont probants. Les résultats aux évaluations d'entrée en sixième des élèves

Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur les difficultés à mobiliser nos territoires pour les jeux Olympiques et Paralympiques prévus à Paris en 2024.

Or, actuellement, une certaine déception se fait sentir, compte tenu notamment d'une communication et d'une implication insuffisantes. Les bonnes volontés sont ainsi découragées, alors qu'elles ne manquent pas, et pas seulement au sein des CDOS. CDOS. On constate ainsi un manque de déclinaison locale de certaines démarches, comme le label « Terre de Jeux 2024 » ou l'absence de conférences animées par des personnalités du monde du sport, même si on comprend que la crise sanitaire ne permette pas les rassemblements habituels. Le label ne semble pas avoir été très attractif pour les collectivités territoriales, et l'on ne peut que déplorer le manque de moyens de communication des structures locales, qui ne peuvent développer leur intérêt dans cette démarche. De même, on constate une véritable difficulté à communiquer auprès des entreprises et à les mobiliser alors qu'elles peuvent constituer des viviers dans les solutions locales dans le cadre d'« Entreprises 2024 ». Nous avons constaté tout cela dans les Ardennes, même si nous comptons treize sites labellisés. nombreuses collectivités locales et entreprises aimeraient pourtant participer à cet effort, qui doit permettre une organisation optimale des jeux Olympiques et leur rayonnement.

Nous avons besoin de retombées locales et du dynamisme de nos territoires.

plus de 1 400 collectivités de tous niveaux- communes, EPCI, départements et régions -ont adhéré à ce programme. Afin d'animer cette communauté, le premier forum

Dans son prolongement, des webinaires ou réunions virtuelles thématiques sont organisés régulièrement afin de permettre un échange direct avec les labellisés « Terre de Jeux 2024 ».

Je rappelle que les labellisés peuvent retrouver l'ensemble de ces informations sur les sites ou dans une mensuelle. Parallèlement, le COJO a également lancé en juin 2019 l'appel à projets sur les Centres de préparation aux jeux ayant vocation à accueillir des délégations étrangères de sportifs de haut niveau en stage de préparation pour les jeux de Paris, entre l'automne 2021 et l'été 2024. Après la clôture des candidatures à la labellisation CPJ, les dossiers ont été instruits par le COJO, avec le concours des services déconcentrés du ministère chargé des sports au premier semestre de 2020. Le 5 octobre 2020, le COJO a annoncé la labellisation de 620 CPJ à travers toute la France. Dans chaque département où au moins une candidature avait été présentée, au moins un centre a été labellisé. Le département des Ardennes, quant à lui, en compte cinq Bogny-sur-Meuse, la salle Reine Bestel à Charleville-Mézières, la maison départementale des sports, le site des Vieilles Forges et le complexe sportif du Bois du Han. De plus, l'État consacrera 20 millions d'euros sur deux ans- en 2021 et en 2022 -au financement de travaux ou d'achats de matériel pour aider les CPJ qui en auraient besoin. Enfin, avant la fin du premier semestre de 2021, une communication institutionnelle sera réalisée auprès de l'ensemble des collectivités concernées. La parole

Ces derniers sont uniques en France et sont occupés par des enseignants spécialisés qui interviennent au plus près des élèves. Ce faisant, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés a presque doublé, et nous nous en félicitons. s'est pas accompagnée d'une hausse proportionnelle du nombre de postes de personnels spécialisés. Lors de la réunion du groupe de travail du 21 janvier 2021, le directeur académique a fait part de son souhait de fermer les 33,5 postes de conseillers et de les transformer d'enseignants référents. Cette suppression signifie la fin des interventions pédagogiques au sein des établissements scolaires : interventions dans les classes auprès des élèves, conseils aux enseignants, formation, prises de poste et accompagnement des AESH, participation aux réunions des directions d'écoles, aide à la constitution des dossiers auprès des MDPH, lesquels nécessitent de nombreux entretiens avec les familles. Cette décision a pu être annulée

en Seine-Saint-Denis. Tout d'abord, les postes de conseillers d'aide à la scolarisation, vous le savez, n'ont pas été supprimés ni transformés en postes d'enseignants référents. Sur le terrain, les autorités académiques structurent un réseau de professionnels pour accompagner les équipes et les élèves. Il est constitué de coordonnateurs, au nombre de 66 en Seine-Saint-Denis ; de conseillers pédagogiques ; de conseillers d'aide à la scolarisation correspondant à 33,5 équivalents temps plein, soit un par circonscription ; d'enseignants référents à hauteur de 36 équivalents temps plein ; d'AESH référents.

Par ailleurs, des AESH référents sont en cours de recrutement pour être des pairs experts dans l'accompagnement de la professionnalisation des AESH, à raison d'un par district, soit huit pour la Seine-Saint-Denis. Enfin, pour renforcer sur le terrain la coopération entre tous les acteurs autour du parcours des enfants, la politique de l'école inclusive est portée par un service départemental organisé pour répondre aux besoins de tous les professionnels et usagers. Le Comité départemental de suivi de l'école inclusive réunit les partenaires- l'ARS, la MDPH,

(JIRS) en Guyane. Il existe actuellement huit JIRS, lesquelles ont été créées par une loi de 2004. Ces juridictions regroupent des magistrats du parquet et de l'instruction qui disposent d'une compétence et d'une expérience particulières en matière de lutte contre la criminalité organisée et de délinquance financière. Leurs moyens techniques renforcés leur permettent ainsi de mener à bien leurs enquêtes, notamment en matière de trafic de stupéfiants et d'infraction commise en bande organisée. Actuellement, la JIRS de Fort-de-France est compétente pour les Antilles et la Guyane. Or, outre que le territoire guyanais se trouve dans le bassin amazonien, dont les spécificités sont totalement différentes de celles du bassin caribéen, la Guyane est désormais confrontée à un trafic exponentiel de stupéfiants en provenance des pays voisins, en particulier du Suriname, et à une montée de la délinquance et de la criminalité liée à ce narcotrafic. La création d'une JIRS amazonienne en Guyane apparaît de plus en plus nécessaire ; celle-ci aurait pour mission de lutter sur le terrain et à l'échelle transfrontalière contre le trafic de stupéfiants, qui détruit la société guyanaise et dont les effets s'exportent vers l'Hexagone, la Guyane étant devenue l'une des grandes portes d'entrée de la cocaïne en Europe. Une telle structure permettrait d'être très efficace sur le terrain, car on déploierait des moyens qui doivent être proportionnels aux défis transfrontaliers qui se posent à notre État au niveau sud-américain. La situation n'est plus la même qu'en 2004. Le rattachement de la Guyane à la JIRS de Fort-de-France est donc désormais totalement inadapté inadapté au regard des mutations survenues dans la grande région amazonienne en termes de trafics transfrontaliers. Le ministère de la justice sait s'adapter en fonction des évolutions. Il l'a prouvé, par exemple en recréant une cour d'appel de plein exercice à Cayenne

ministre déléguée. Madame la sénatrice, comme vous l'avez parfaitement rappelé, la Guyane, département frontalier du Brésil et du Suriname, est située dans le ressort de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, compétente pour connaître d'affaires de criminalité organisée et financière de grande complexité, tant dans les Caraïbes qu'en Guyane. Cette organisation se traduit par une prise en charge effective de la délinquance organisée guyanaise, notamment le narcotrafic, dont vous dénoncez à juste titre les ravages.

Très concrètement, vous avez raison : le nombre d'affaires de Guyane suivies par la JIRS de Fort-de-France a nettement augmenté depuis 2004. Le nombre total de dossiers guyanais traités ou en cours de traitement par cette juridiction depuis 2004 s'élève au nombre de

Le nombre de dossiers en provenance de la Guyane donnant lieu à saisine de la juridiction est passé d'une moyenne de 1,25 entre 2004 et 2017 à une moyenne de 4,3 au cours de la période 2018-2020. Cette évolution de la délinquance apparaît toutefois correctement prise en charge à ce stade par la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, qui a su s'adapter aux défis que connaît la Guyane en matière de criminalité organisée. la Guyane bénéficie de l'expertise spécifique et des moyens, renforcés depuis 2019, de la JIRS de Fort-de-France- affectation supplémentaire d'un magistrat du parquet, d'un juge d'instruction et d'un assistant spécialisé douanier définit sa politique pénale en prenant précisément en compte les spécificités de la criminalité organisée guyanaise et en s'attachant à renforcer la coopération internationale sur la zone, grâce, notamment, à l'appui du magistrat de liaison basé au Brésil, compétent sur le Suriname. Enfin, le périmètre de compétence d'une juridiction interrégionale spécialisée s'inscrit, par construction, sur un espace interrégional. Une création se limitant au seul département de la Guyane serait donc contradictoire avec l'objet même de cette organisation judiciaire, qui vise à mutualiser les moyens en donnant une taille critique au ressort au ressort de chaque juridiction afin d'en améliorer l'efficacité. Pour toutes ces raisons, il n'est pas, à ce stade, envisagé de créer une telle juridiction spécifique en Guyane, qui viendrait amoindrir la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, laquelle est compétente en Guyane et dans les Antilles françaises. Toutefois, vous le savez,

La crise sanitaire a eu et a encore un effet ciseau pour ces collectivités : une forte baisse des recettes touristiques et une augmentation des dépenses, notamment liées au soutien à l'économie locale.

Rallonger la durée des travaux ou en réduire le nombre est particulièrement dommageable pour le tissu économique local et français dans son ensemble, notamment pour les entreprises du BTP, qui ont besoin de la commande publique. Cela est tout particulièrement préjudiciable pour des communes qui se battent au quotidien pour rester attractives sur les marchés nationaux et internationaux. Il serait donc opportun de prévoir une exception comptable afin que les communes puissent étaler les dépenses liées à la crise sanitaire sans avoir à rogner sur des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Aussi, madame la ministre, pourriez-vous nous préciser quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour permettre aux collectivités territoriales, en particulier aux communes touristiques comme celles du golfe de Saint-Tropez, de lisser, peut-être sur plusieurs années, leurs dépenses liées à la covid-19 et ne pas mettre en péril leurs investissements, si essentiels pour l'attractivité de leurs territoires et de la France en général ? ministre déléguée. Madame la sénatrice Dumont, votre question porte sur les difficultés financières rencontrées par les communes touristiques, en particulier par celles du golfe de Saint-Tropez, dans le Var, dans le contexte de la présente crise sanitaire. sanitaire. Je tiens tout d'abord à rappeler les engagements pris par le Gouvernement pour faire face, grâce à de multiples dispositifs de soutien, aux conséquences de cette crise, tant pour les acteurs de la sphère privée que pour ceux de la sphère publique. et des relations avec les collectivités territoriales, le ministère de l'économie, des finances et de la relance s'est tout particulièrement mobilisé, depuis le printemps 2020, pour accompagner les collectivités locales dans la gestion de cette crise sanitaire sans précédent. Au-delà du nécessaire assouplissement du calendrier de reddition des comptes de l'exercice 2019, les conditions de l'équilibre des budgets des collectivités locales ont été, comme vous le soulignez à juste titre, au coeur des préoccupations du Gouvernement, tout au long de l'année 2020, et le sont encore, naturellement, en 2021. Cette mobilisation s'est tout d'abord traduite par la mise en oeuvre de dispositifs visant à garantir, sous certaines conditions, le niveau des ressources allouées aux collectivités locales. Les pertes liées à l'activité touristique font ainsi l'objet d'une attention particulière dans le dispositif de garantie des recettes communales prévu à l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020. En effet, les pertes liées à la baisse des recettes de taxe de séjour sont prises en compte, et dans des conditions plus favorables que les autres taxes figurant dans le panier de recettes, car la perte de taxe de séjour est estimée par rapport aux recettes de la seule année 2019 et non par rapport à la moyenne des recettes des années 2017, 2018 et 2019. Cette garantie a été reconduite en 2021, comme vous le savez, par l'article 74 de la loi de finances pour 2021, avec la même référence à l'année 2019. Par ailleurs, le traitement budgétaire et comptable des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du covid-19 a fait l'objet d'une attention toute particulière. Ainsi, la circulaire interministérielle du 24 août 2020 a prévu des mesures spécifiques d'adaptation du cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette circulaire vise à préserver les équilibres budgétaires tout en assurant la traçabilité des dépenses mobilisées pour faire face à la crise. À cet égard, et pour répondre à votre demande et à celle des collectivités locales, les dépenses engagées par les collectivités locales peuvent être étalées sur une durée maximale de cinq ans. Parmi les dépenses concernées, on peut citer les dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire, le soutien au tissu économique, dès lors que les règles de compétence et de marchés publics sont respectées, ou encore les subventions d'équilibre aux budgets annexes, ainsi que les subventions, contributions ou participations à différentes structures résultant des effets de la crise sanitaire. Il faut conclure ! Ces mesures budgétaires et comptables dérogatoires ont été étendues par circulaire interministérielle du 15 février 2021 aux dépenses engagées au cours du premier semestre de 2021. Enfin, je tiens à souligner que la mise en oeuvre de ces mesures s'est inscrite dans le cadre d'une étroite concertation avec les représentants des associations d'élus. Vous pouvez compter sur le Gouvernement pour continuer de suivre de très près cette situation.

de la relance. Je souhaite interroger le Gouvernement sur la présence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sur la liste des organismes divers d'administration centrale, dits ODAC, ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois. L'inscription de l'AEFE sur cette liste l'empêche d'accompagner la croissance du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger, alors que celui-ci prévoit de doubler le nombre des élèves qu'il scolarise De nombreux établissements scolaires en gestion directe sont bloqués dans leurs projets immobiliers, faute pour l'AEFE d'une capacité d'emprunt. Pourtant, ces EGD sont largement financés par les frais de scolarité payés par les familles ; les emprunts qui pourraient être contractés seraient donc remboursés grâce à l'augmentation des recettes engendrée

très vite remboursé. L'attribution de cette capacité d'emprunt a été demandée par le directeur de l'AEFE lors d'un comité interministériel en janvier 2021. Elle faisait aussi partie des principales recommandations du rapport conjoint des inspections des affaires étrangères et de l'éducation nationale remis au Gouvernement au printemps 2019. Ce rapport rappelait d'ailleurs que plusieurs établissements publics avaient été radiés de la liste des ODAC, comme Mines ParisTech, le CNED ou l'IGN. Il convient aussi de constater que la subvention publique est de plus en plus minoritaire dans les recettes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. En effet, ses ressources propres, qui proviennent, d'une part, des frais de scolarité payés par les familles dans les établissements en gestion directe et, d'autre part, de la facturation des personnels et des services rendus aux établissements conventionnés, sont en constante augmentation depuis plusieurs années. plusieurs années. Le Gouvernement envisage-t-il vraiment de donner à l'AEFE la capacité de participer à la croissance du réseau de l'enseignement français à l'étranger ? ministre déléguée. Monsieur le sénateur Leconte, vous m'interrogez sur l'inscription de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sur la liste des organismes divers d'administration centrale, les fameux ODAC, qui ne l'autorise pas à s'endetter auprès d'un établissement de crédit sur une durée supérieure à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excéderait cette durée. Cette interdiction, décidée par le législateur, vise à mieux maîtriser la dette publique et les dépenses associées à sa charge et à mieux maîtriser la dissémination de l'endettement public entre les différents organismes. La qualification en ODAC est établie tous les ans par l'Insee de manière indépendante suite d'une étude approfondie de chaque entité. Cela ne se décrète donc pas. Plusieurs critères sont pris en compte lors de cette étude, tels que le poids de l'État dans la gouvernance et les modalités de financement de l'organisme, en particulier sa part respective des ressources propres et des financements publics. Ces éléments sont pris en compte de manière globale. Une seule variation ne conduit pas à remettre en question cette classification. Le ministère chargé des comptes publics adopte un arrêté qui ne fait que reprendre, en pratique, les classifications opérées par le comptable national. C'est une question de crédibilité, notamment à l'endroit de nos financeurs. Toutefois, l'attention de l'Insee pourra être attirée sur une éventuelle révision de la qualification de l'AEFE, décidée chaque année. Toute évolution ne pourra résulter que de changements significatifs et objectifs dans le modèle économique de l'AEFE par rapport à la situation antérieure qui avait conduit à sa qualification en ODAC. Indépendamment d'une éventuelle requalification, des solutions substitutives à l'endettement, qui reposeraient en particulier sur la trésorerie abondante de l'AEFE, peuvent être mises en oeuvre pour répondre à l'objectif, parfaitement légitime, de lui donner les moyens de son développement. trésorerie atteint, en 2020, environ 300 millions d'euros, dont environ 150 millions d'euros pour les établissements en gestion directe. Mis en commun, ces montants permettraient d'absorber largement les besoins d'investissement immobilier du réseau de ces établissements en gestion directe. Le nouveau contrat d'objectifs et de moyens, en cours d'élaboration, doit être l'occasion de normaliser les modalités de financement de l'immobilier des établissements en gestion directe en mettant fin aux avances dérogatoires de l'Agence France Trésor et en actant une évolution dans le sens d'une mise en commun

Depuis le décret du 29 octobre 2020, leurs espaces de salon de thé sont à nouveau fermés, au même titre que les restaurants, ce qui représente une perte de plus de 70 % de leur chiffre d'affaires. Or ces entreprises ne perçoivent aucune aide sur la partie salon de thé. Par une question écrite en décembre dernier, puis par un courrier en date du 25 janvier, resté malheureusement sans réponse à ce jour, j'avais déjà alerté le Gouvernement sur cette situation. J'associe à cette question orale mon collègue du Haut-Rhin, le sénateur Christian Klinger, qui a, lui aussi, été interpellé à ce sujet dans son département. En Alsace, les salons de thé-pâtisseries font partie de notre tradition. Nous y sommes fortement attachés. À l'heure actuelle, leurs pertes financières s'élèveraient à 170 000 euros ; qui plus est, disposer d'un espace de salon de thé en plus de la surface de vente conduit à payer un loyer et des charges plus importants. Des pâtisseries-salons de thé craignent de devoir licencier ou fermer. Je me fais ici l'écho du président de la chambre de métiers d'Alsace : « Si l'on ne fait rien, ces entreprises, symbole de notre art de vivre alsacien, vont tout simplement disparaître. Depuis un an, les salons de thé-pâtisseries demandent à bénéficier des mêmes aides que les restaurateurs. Certes, des aides économiques existent, mais ces dispositifs ne tiennent pas compte de l'activité de salon de de salon de thé. J'ai notamment pu échanger avec les gérants d'une pâtisserie strasbourgeoise, qui m'ont indiqué perdre de l'argent à chaque fois qu'ils ouvraient leur commerce. Il est urgent entendre et de répondre à cette forte inquiétude, relayée par toute une profession, et d'apporter une lueur d'espoir, dans ce contexte ô combien compliqué, aux 400 professionnels alsaciens qui correspondent à ce cas de figure. Madame la ministre, comment comptez-vous prendre en compte cette situation particulière- ô combien importante ! -des salons de thé-pâtisseries-boulangeries ? La parole ministre déléguée. Madame la sénatrice Schalck, vous appelez mon attention sur la situation des entreprises multi-activités, notamment sur celle des pâtisseries-salons de thé, qui réalisent 75 % de leur chiffre d'affaires grâce au salon de thé. Au titre de l'aide du mois de février 2021, toutes les entreprises, quels que soient leur chiffre d'affaires et leur secteur d'activité, sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité. Aujourd'hui, l'activité principale détermine le régime d'aide dont peut bénéficier une entreprise ayant plusieurs activités, définie comme celle qui contribue le plus au chiffre d'affaires de référence, indépendamment du code NAF de l'entreprise. Pour calculer le montant de l'aide, la perte de chiffre d'affaires est déterminée à partir du chiffre d'affaires de référence, toutes activités confondues. Prenons le cas d'une pâtisserie-salon de thé

En revanche, si le principal chiffre d'affaires est réalisé par l'activité de pâtisserie, qui continue de fonctionner, l'entreprise pourra néanmoins bénéficier du régime d'aide des entreprises des secteurs dits S1 dont la pâtisserie fait partie, conformément à l'annexe 2 du décret relatif au fonds de solidarité. Toutefois, si les conditions d'accès au fonds de solidarité sont différentes pour ces deux régimes d'aide- les entreprises des secteurs S1 subir une perte de plus de 50 % de leur chiffre d'affaires, ainsi qu'une perte de 10 % sur l'année 2020 -, les niveaux d'aide pour ces deux régimes sont désormais quasiment alignés. Là encore,

disposition législative ne permet d'établir une distinction entre les personnes valides et celles qui présentent un handicap ou une invalidité pour l'accès aux prêts et aux crédits bancaires, nous savons que, dans les faits, la situation est tout autre.

en réalité, les personnes en situation de handicap, plus encore celles qui bénéficient de l'AAH (allocation aux adultes handicapés), ont toutes les peines du monde à obtenir des prêts. Les difficultés sont principalement de deux ordres. Les banques ou organismes de crédit prêtent sur la base de l'examen des ressources et des revenus et ne considèrent pas l'AAH comme un revenu. Certains justifient même leur refus par l'interdiction qui leur est faite de prêter à quelqu'un d'insolvable. Or l'AAH étant, en principe, insaisissable, la personne qui la perçoit est considérée comme telle. Lorsque les revenus ne sont pas un obstacle, c'est le questionnaire médical qui discrimine, par le biais de l'impossibilité de trouver une assurance emprunteur. La convention Aeras- s'assurer et emprunter

d'assurance proposées à une jeune femme en situation de handicap pour un prêt immobilier supérieur à 320 000 euros avaient été fixées à 1 500 euros par mois ! Ces difficultés conduisent bien souvent les personnes en situation de handicap à s'orienter vers des solutions spécifiques et à portée limitée- CAF, courtiers ou organismes spécialisés, prêts entre particuliers -ou, tout simplement, à renoncer au crédit. Il s'agit d'une discrimination masquée qui ne dit pas son nom, mais qui est bien réelle. D'ailleurs, lorsque celle-ci peut être prouvée, les actions en justice donnent systématiquement raison aux personnes discriminées, sans que cela leur ouvre droit à un emprunt pour autant.

Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Gréaume, je tiens avant tout à vous assurer du plein engagement du Gouvernement pour assurer aux personnes en situation de handicap un accès équitable au crédit bancaire. Toute discrimination des personnes en situation de handicap

Toutefois, au regard des remontées dont nous disposons et au-delà de quelques cas regrettables qui peuvent survenir et contre lesquels nous devons agir fermement, nous ne constatons pas de blocage généralisé pour l'accès au crédit bancaire des personnes en situation de handicap. comme vous le rappelez, des mécanismes existent, tels que la convention Aeras- s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé -, qui permet aux publics concernés de bénéficier d'un examen spécifique de la demande d'assurance et d'un plafonnement des cotisations d'assurance emprunteur. Cette convention, qui permet de limiter la charge d'assurance et donc de faciliter l'accès au crédit, fonctionne de manière satisfaisante et a été renouvelée en 2020. L'ensemble de ces dispositions a pour objectif d'assurer un meilleur accès au crédit pour les personnes avec un risque de santé aggravé.

que nombre d'enquêtes montrent que celles-ci sont déjà particulièrement impactées par la situation économique et sociale. Il y a urgence à agir contre ceux qui n'autorisent pas les emprunts.